Le code général des impôts prévoit le remboursement des accises à l'opérateur professionnel qui a expédié des produits pour lesquels les droits d'accise ont déjà été acquittés.

le plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d'aménagement du territoire qui lui est confiée. Ces abattements viennent alimenter le Fonds postal national de péréquation territoriale. Ce fonds contribue au maintien de services postaux sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements et régions d'outre-mer. Il contribue également au financement financement des maisons de services au public et des futures maisons France Service hébergées par La Poste. Compte tenu de la diminution de l'allégement fiscal prévu à l'article 1635 du code général des impôts consécutive à l'érosion de la valeur ajoutée qui constitue la base d'imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le relèvement du plafond actuel, de 95 % à 99 %, permettra de garantir la stabilisation de la compensation par l'État de cette mission de service public à hauteur de 174 millions d'euros par an. Le produit des impositions directes locales de La Poste étant affecté à l'État, cette mesure impacterait les recettes du budget général. Mes chers collègues, je

par Poste Immo et ses filiales, afin de financer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste. Ces abattements viennent alimenter le Fonds postal national de péréquation territoriale. Ce fonds contribue au maintien de services postaux sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d'outre-mer. Il contribue également au financement des maisons de services au public et des futures maisons France Service hébergées par La Poste. Afin de renforcer le financement de cette mission, qui correspond à une attente forte des populations sur les territoires, il est proposé, dans le cadre de la préparation du prochain contrat de présence postale territoriale 2020-2022 entre l'État, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité et La Poste, d'instaurer une ressource supplémentaire supportée par les collectivités locales. Cette ressource proviendra d'un allégement des taxes foncières dues par les foncières de La Poste, filiales de Poste Immo, pour les immeubles qui sont affectés à titre principal ou exclusif aux activités de La Poste. Cet allégement sera plafonné à 10 et calculé sur la base de la valeur des immeubles dans lesquels s'effectue l'activité du service postal. Cette mesure permettra de dégager un financement de l'ordre de 3 millions d'euros par an. Elle sera

activité. En l'état de la législation, un entrepreneur assujetti à l'impôt sur le revenu doit l'acquitter sur l'intégralité du bénéfice, y compris sur la part qu'il décide de réinvestir dans l'entreprise

tend à prévoir que, « lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, cette exonération s'applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l'ensemble de ces entreprises

Cet amendement vise à rétablir un peu de justice fiscale entre tous les acteurs du commerce. En 2018, la fiscalité sur le commerce physique a rapporté 47,3 milliards d'euros, générés par près de 90 impôts, parmi lesquels 26 taxes contribuant à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, alors qu'ils sont en pleine croissance économique, les géants du numérique ne sont pas soumis aux mêmes règles d'équité. La contribution fiscale des GAFA au titre du commerce physique n'a représenté que 67 millions d'euros. Le commerce électronique bénéficie d'une fiscalité allégée du fait de son mode de fonctionnement et d'organisation. En particulier, les acteurs économiques « qui ont des entrepôts de stockage n'étant pas intégrés à des magasins de commerce de détail profitent pleinement de l'espace public sans pour autant contribuer aux charges de celui-ci.

Parce qu'ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu'ils réalisent une véritable opération de vente commerciale, à l'image des magasins

sols. Ces surfaces de stockage consomment trois fois plus d'espace que la distribution physique traditionnelle. L'objet de cet amendement est donc d'internaliser le coût environnemental de l'artificialisation des sols induite par la construction de ces nouveaux centres logistiques et de stockage. Pour lutter contre cette artificialisation, il convient, sans créer de nouvelles taxes, de supprimer les incohérences législatives incitant à la consommation d'espace. Allons-nous rester spectateurs de ces destructions ? Car il s'agit bien de destructions ! Une surface artificialisée est une surface morte, et ce pour longtemps.

d'imposer des choix aux consommateurs. En revanche, la responsabilité du législateur d'un point de vue fiscal est d'assurer une équité de traitement. C'est ce que nous avons fait-

La parole est à M. le rapporteur général,

concerne les nouveaux établissements de stockage et de logistique dont les permis de construire ont été délivrés après le 1 juin 2020 et qui devraient servir à la vente de biens à distance.

centres-villes. Il vise à moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces. Si l'établissement se situe en centre-ville, le montant de la taxe est réduit de 50 % alors qu'il est majoré de 50 % si le commerce se situe hors centre-ville, hors centre-ville, c'est-à-dire en périphérie. L'objectif est de privilégier l'implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu'en périphérie.

des grandes surfaces en intra-urbain, qu'il convient d'accompagner. La modulation d'une taxe existante comme la Tascom permettrait d'agir en faveur de la revitalisation des centres-villes.

Cet amendement vise à favoriser les commerces de villes et de centres-bourgs, conformément aux engagements du Gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé « Action coeur de ville ». À cette fin, il est proposé de moduler progressivement le taux de la taxe sur les surfaces commerciales selon le lieu d'implantation des grandes surfaces, dans une logique de « bonus-malus ». Il tend également à introduire une majoration additionnelle progressive au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d'établissements concernés par la Tascom, hors villes et centres-bourgs, à partir du 1 juin 2020. L'objectif est de privilégier l'implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu'en périurbain, où l'implantation commerciale a souvent les multiples conséquences que j'ai évoquées précédemment. Le bonus que tend à prévoir cet amendement est de nature à réduire le coût d'exploitation des commerces de centres-villes et de centres-bourgs,

un avis défavorable

de la taxe sur les surfaces commerciales. L'objectif de cette majoration était de compenser les avantages de la mise en place du CICE- nous avons vu qu'ils étaient discutables -perçus par la grande distribution alimentaire et non alimentaire. Le CICE a été transformé en allégements de charges et réduit

Le produit de cette majoration serait affecté à l'État. Cette majoration s'inscrit dans le droit fil des majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 réalisant un chiffre d'affaires de plus de 3 000 euros par mètre carré, et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L'amendement vise donc à permettre de taxer davantage les grandes surfaces commerciales,

à promouvoir une économie et des commerces de proximité, et à défendre les centres-villes. La désertification des centres, dans les petites villes et les villes moyennes, est en effet un sujet qui nous concerne tous. Les amendements

les confréries constituées en associations, qui contribuent au rayonnement culturel, patrimonial et touristique de leurs régions. Pour ce faire, ces confréries doivent répondre à une double condition

puisqu'il permet de ne pas imposer les bénéfices des organismes dont la gestion est désintéressée, sous réserve que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante et que le montant de leurs recettes annuelles correspondant aux activités lucratives n'excède pas 63 059 euros, seuil

de reconversion de friches industrielles ou commerciales que vous visez, monsieur le sénateur, peuvent d'ores et déjà bénéficier de ce dispositif lorsqu'elles sont situées dans des zones tendues en matière de logement. Votre amendement a pour objet d'inciter à la reconversion de friches en logements dans des zones non tendues,

Je ferai un parallèle avec l'article 7 proposé par le Gouvernement, qui prévoit la limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d'en garantir l'évaluation. Notre amendement entre tout à fait dans ce dispositif Cette niche existe depuis 2005 : il serait peut-être temps de la limiter. La parole

Le CPO estime qu'elle correspond parfaitement « à l'objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l'attrait d'un certain nombre d'opérations en capital ». C'est un avis positif. Dès lors, nous ne souhaitons pas

dans les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) passent d'un régime réel d'imposition à un régime de micro-entreprise, ou inversement. inversement. S'agissant des bénéfices agricoles, en cas de passage d'un régime réel au régime « micro-BA », les recettes du premier exercice d'application du régime micro-BA seraient diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel. En effet, ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d'imposition. Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 de permettre la déduction des charges correspondantes. La même logique s'applique aux bénéfices non commerciaux. L'amendement tend à insérer cet article additionnel d'avancer au 1 janvier 2020 l'entrée en vigueur de ces dispositions, laquelle était initialement prévue au 1 janvier 2021.

L'article 15 prévoit une baisse de 380 millions d'euros d'ici à 2023 de la taxe pour frais de chambre, dont 80 millions d'euros en 2020. Le groupe socialiste s'était opposé, lors de l'examen de la loi Pacte, à la réforme qui impacte fortement l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Nous étions notamment opposés aux mesures qui visent au développement de l'activité des CCI dans le champ concurrentiel et à l'obligation de recrutement de salariés de droit privé.

prévue dans le contrat d'objectifs et de performance qu'il a signé avec les CCI en avril dernier. Par ailleurs, cette trajectoire budgétaire impactera avant tout les CCI rurales,

dont la survie est menacée par un tel niveau d'économies. L'instauration d'une clause de revoyure permettrait aux différentes parties de tirer de premières conclusions sur cet effort budgétaire et

entre CCI France et le ministre de l'économie et des finances. Du fait de la trajectoire à la baisse des ressources du réseau des CCI, il y a lieu de prévoir une concertation afin de prendre en compte les obligations du réseau au regard des moyens mis à sa disposition.

et des finances le 15 avril 2019 prévoit une clause de revoyure annuelle afin d'étudier spécifiquement la soutenabilité pour le réseau des CCI de la trajectoire de sa taxe affectée.

afin d'adapter, si nécessaire, le dispositif d'ensemble, et notamment l'évolution du plafond de la taxe affectée, au regard des impacts économiques, sociaux et territoriaux observés, incluant la capacité pour les CCI de mobiliser des co-financements et d'augmenter le volume de facturation. La taxe pour frais de CCI étant soumise, comme toutes les taxes, au contrôle du Parlement, la formalisation de cette clause de revoyure sous la forme d'un rapport annuel rédigé par CCI France et remis à son ministre de tutelle est souhaitable. Cet échange formel, sanctuarisé dans la loi,

Par ailleurs, le mécanisme proposé ne nous paraît pas le plus approprié pour assurer une répartition des ressources adaptées aux besoins de chaque chambre : d'une part, des CCI peuvent être en difficulté en dehors des zones très rurales,

Pour autant, il ne nous paraît pas opportun de baisser de moitié le taux de cette taxe au motif que le taux d'intérêt de retard a lui-même baissé de moitié au 1 janvier 2018. cette taxe n'a pas seulement pour objet de réparer le coût du temps supporté par l'État du fait de la perception différée de sa créance. Elle a aussi une vertu dissuasive : il s'agit d'inciter les entreprises d'assurances à faire preuve d'une plus grande rigueur dans la constitution de leurs provisions fiscalement déductibles et de les dissuader de sur-provisionner

Nous avons dû le réclamer à maintes reprises, pour qu'il nous soit envoyé lundi après-midi. Or, objectivement, avec les seules réponses aux questionnaires budgétaires et une consultation du site du Grand Paris, nous aurions pu rédiger exactement le même rapport ... Ce document ne

Nous souhaitons qu'une solution alternative pérenne et plus équilibrée soit trouvée pour éviter cette augmentation systématique de la taxe sur les bureaux, tout en garantissant le financement du Grand Paris Express. La

perdition, en tout cas budgétaire, on ne s'y prendrait pas autrement ! La question à laquelle il faudrait que le Gouvernement réponde, c'est : où en est-on du coût réel de ce projet ?

Je pense néanmoins que si le Gouvernement souhaite des recettes, c'est probablement qu'il y a eu des dépassements importants et que cet argent est nécessaire. Je ne pense pas que ce soit par plaisir de créer des taxes nouvelles

vous voyez bien que l'offre est nettement inférieure à la demande en matière de bureaux et d'installation d'activités économiques. On ne fait donc pas peser

Il est notamment fait l'hypothèse que la SGP percevra de l'ordre de 1,35 milliard d'euros de recettes nettes en 2031. Ce chiffre repose sur une hypothèse de travail supposant des recettes complémentaires augmentant progressivement

Les hypothèses retenues seront vérifiées annuellement dans le cadre des éditions successives de ce rapport, de manière à ajuster éventuellement les ressources affectées et à garantir la soutenabilité du modèle. »

clairement le rôle des collectivités territoriales face à la tutelle de l'État, qui ne perd jamais une occasion d'affaiblir l'attractivité économique de la capitale et de sa région.

Cet amendement a pour objet de remettre à la charge de l'État le coût de l'allégement de la taxe d'habitation prévu pour 2019 en faveur des contribuables qui bénéficiaient déjà en 2018 du dispositif de sortie en sifflet.

reprend en matière de compensation exactement les dispositions adoptées en 2017 et en 2018-il y a donc une forme de continuité. Nous avons modifié l'équilibre budgétaire afférent à hauteur de 226 ou 227 millions d'euros.

L'application d'un droit fixe de 125 euros est dérogatoire au régime de droit commun des droits de mutation. Elle est conçue pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs et particuliers, notamment dans un cadre familial. Il nous paraît inopportun, pour ne pas dire contradictoire, de subordonner la mise en place ou le maintien de régimes fiscaux dérogatoires en anticipant des hypothèses d'optimisation, et ce d'autant plus que nous n'avons pas connaissance d'opérations d'optimisation autour d'un montant de 125 euros. Les conditions prévues ne permettent pas d'atteindre l'objectif souhaité par les auteurs de l'amendement. Certaines de ces conditions sont insuffisamment précises- comme le cahier des charges d'au moins dix ans sans détail sur le contenu -, et incohérentes avec le risque évoqué d'opérations spéculatives de plusieurs millions d'euros si la valeur de cession est inférieure à 250 000 euros, l'écart étant majeur.

L'amendement n° I-272 rectifié n'est pas soutenu. Quel est l'avis de la commission

Il convient donc de faciliter les échanges permettant d'opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l'exploitation en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d'immeubles ruraux ne sont applicables qu'à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes du canton. Cette limitation géographique pour le moins paradoxale est aujourd'hui difficilement justifiable justifiable dans la mesure où l'échange est d'autant plus bénéfique qu'il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d'une parcelle proche du centre de l'exploitation. C'est pourquoi il est proposé de supprimer les conditions de proximité géographique pour l'application des dispositifs de faveur aux opérations d'échanges d'immeubles ruraux. En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. compte tenu de la fiscalité applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.

des échanges d'immeubles ruraux, quel que soit l'emplacement géographique des biens échangés, et quelle que puisse être la finalité de l'échange des biens situés hors du même canton ou des communes limitrophes. Il n'y aurait donc aucun ciblage,

L'Inspection générale des finances, dans un rapport de 2014, avait répertorié 192 taxes à faible rendement. Dans cet article, vous proposez, monsieur le secrétaire d'État, d'en supprimer 18. Comme l'a bien analysé le rapporteur général, certaines suppressions vont de soi lorsqu'elles concernent les recettes de l'État et lorsqu'il s'agit de mesures de simplification du droit fiscal, certaines taxes ayant un rendement quasi nul et un coût de recouvrement disproportionné.

Par ailleurs, dès lors que l'État n'est pas impacté et qu'il s'agit parfois de ressources des collectivités locales, pourquoi les remettre en cause alors qu'aucun débat, notamment avec le Comité des finances locales, n'a eu lieu

Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts doivent acquitter, au profit des communes et des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite. Le montant de cette redevance est fixé respectivement à 2 et 3,5 euros de production. Ce dispositif, instauré par l'article 138 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi

Ces dispositions ne sont cependant jamais entrées en vigueur en l'absence de la publication, par le Conseil d'État, d'un décret, pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La suppression de cette redevance serait préjudiciable à la commune de Bouillante et à la région de Guadeloupe. En se basant sur la production de 2017, le montant des recettes générées en application de l'article 138 de la loi ÉROM s'élèverait chaque année à 230 000 euros pour la commune de Bouillante et à 395 000 euros pour le conseil régional de Guadeloupe.

Aussi, le dispositif que nous proposons est plus avantageux pour le théâtre privé que la disposition fiscale que vous souhaitez rétablir. Par ailleurs, le ministère de la culture